donc prêts, si on leur impose un contrat d'engagement républicain- dont on ignore le contenu à ce stade, ce qui est problématique -, à assumer des missions extrasportives. Évitons néanmoins de les submerger de contraintes, de surréglementations ou de tracasseries administratives. Nous sommes en effet

actualisons rapidement le guide de la laïcité dans le sport, afin de leur fournir des indicateurs concrets pour les aider au quotidien. La parole est à M. Michel Savin,

Le rapport de notre collègue Jacqueline Eustache-Brinio l'a parfaitement illustrée, et je pense que nous partageons tous l'idée selon laquelle il convient de renforcer certains contrôles. toutefois important de rappeler que la très grande majorité des clubs sportifs et des associations ne sont pas concernés par le phénomène de la radicalisation islamique. C'est une certitude, mais il ne faut pas pour autant nier la réalité : il est urgent et nécessaire de lutter efficacement et directement contre des dérives qui existent au quotidien et qui ne cessent de prendre de l'ampleur. Des données objectives existent, qui sont désormais très largement documentées. L'article 25 ambitionne de renforcer cette lutte. Pourquoi pas ? Je tiens à saluer le fait qu'il vient également renforcer la protection de l'intégrité physique et morale des pratiquants, notamment des mineurs.

proposé un amendement qui vise notamment à renforcer le contrôle des salles privées. Nous devons faire preuve de lucidité et ne pas nous limiter à des seuls discours d'apparence.

Le sport m'a ouvert les portes des promesses de notre République, ces promesses qui font aussi l'objet de cette loi que vous examinez. Les promesses de la République, c'est l'égalité des chances, la liberté de choix et la fraternité. Depuis mon arrivée au ministère, je défends une vision selon laquelle le rôle central du sport est de faire Nation, d'offrir aux jeunes, parfois fragilisés socialement ou en recherche d'identité et d'idéaux, un cadre sécurisé pour leur épanouissement. Nos clubs sportifs sont des lieux où la citoyenneté se vit et se construit, où tous les citoyens, quels que soient leur origine et leur parcours de vie, se rencontrent et apprennent à se comprendre dans leurs différences, à se tolérer, à se respecter, et à intégrer les règles qui constituent le contrat social qui nous rassemble. Je suis très honorée d'échanger avec vous sur l'article 25 de cette loi. Cet article, que j'ai souhaité, incarne la mobilisation du monde sportif en faveur de la promotion des valeurs de la République et du principe de laïcité. de laïcité. Il donnera au mouvement sportif la possibilité de valoriser, comme vous l'avez dit, ce qu'il fait déjà pour la République et ce qu'il peut faire encore davantage, en lien resserré avec l'État. À travers le contrat d'engagement républicain, qui implique les associations locales, et le contrat de délégation, qui matérialise un niveau supérieur d'engagement pour les fédérations délégataires, nos structures participeront à la promotion des principes de la République, au travers non seulement de plans d'action précis, travaillés avec le ministère des sports, mais aussi d'indicateurs quantifiables et de modalités de restitution.

du sport. Cette réforme engage aussi mon ministère en faveur d'un accompagnement plus qualitatif. En complément des outils de prévention et de sensibilisation qui sont élaborés au niveau interministériel

(CIPDR), nous allons mieux former, pour mieux observer et détecter et, le cas échéant, pour signaler aux autorités judiciaires et administratives les situations potentielles de dérive de radicalisation religieuse ou de dérive communautaire. Au coeur de notre République laïque, ma responsabilité politique est double. Elle consiste d'abord à garantir la liberté de conscience, y compris religieuse, à toutes les pratiquantes et pratiquants du sport sans qu'ils soient ni discriminés ni exclus en raison de l'expression de cette liberté. Ensuite, il relève de ma responsabilité de mener sans faiblesse et sans ambiguïté une lutte contre toute tentative de propagande à l'égard de jeunes vulnérables, une lutte contre toutes les haines et contre les phénomènes de radicalisation. Ces phénomènes sont complexes et j'ai toujours pris soin de ne céder ni aux raccourcis ni au cynisme, en veillant notamment à ne pas confondre le port d'un vêtement avec un acte de prosélytisme. Parallèlement, je serai intransigeante sur le fait qu'aucun comportement de propagande religieuse ou politique ne doit avoir sa place sur un terrain de sport. Pour documenter cette complexité, nous avons engagé des travaux de recherche auprès de l'Institut des hautes études du ministère de l'intérieur. Nous avons aussi confié une mission à l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche. Dans les quartiers prioritaires de la ville, mon action porte sur la mixité des pratiques, dès le plus jeune âge. Les financements de l'Agence nationale du sport sont prioritairement ciblés sur des équipements de proximité et des aides à l'emploi d'éducateur. J'ai également obtenu des moyens inédits lors du dernier comité interministériel à la ville, sous la forme d'aides spécifiques supplémentaires de 36 millions d'euros, pour diversifier l'offre associative dans ces quartiers prioritaires. Ces aides serviront notamment à ouvrir les 1 000 nouveaux terrains de sport de proximité Le sport est notre bien commun. Il se situe à la croisée de toutes nos politiques en matière d'éducation, de santé et de vie en société. Cette richesse plurielle est l'héritage que je souhaite laisser aux générations futures.

Mme Raymonde Poncet Monge. Nous arrivons à l'examen de l'article 25, le premier de la section concernant le sport. Cet article vient entamer la confiance des milliers de bénévoles ou professionnels qui font vivre la promesse républicaine au quotidien. ses dispositions modifient en profondeur le régime de l'agrément pour les fédérations et associations sportives, ainsi que celui de la délégation. Madame la ministre, dans la lignée de l'article 6, vous instaurez le contrat d'engagement républicain comme une des conditions d'agrément pour les 200 000 associations sportives de notre pays. Contrairement à ce qui a été affirmé, la semaine dernière, sur ces travées, le Gouvernement ne le fait pas avec le soutien des associations, puisque le mouvement associatif, qui représente une association sur deux en France, est défavorable à ce contrat. La Défenseure des droits et la Commission nationale consultative des droits de l'homme Jeudi dernier, M. le questeur Philippe Bas a très bien résumé ce qu'était ce contrat d'engagement républicain, en le définissant comme « un coup d'épée dans l'eau, une illusion que toutes les associations signeront ». Il ajoute : « Et après ? » Nous partageons ces propos.

républicain jette la suspicion sur des centaines de bénévoles, présidents de club et éducateurs. Si des dérives existent dans les clubs, elles doivent être combattues et nous disposons déjà d'un arsenal pour le faire. L'instauration d'un agrément à durée limitée est un changement majeur pour les fédérations sportives. Pourtant, des motifs de retrait d'agrément ont déjà été définis et utilisés, lorsque c'était nécessaire. Vous souhaitez également que les fédérations délégataires établissent une stratégie nationale visant à promouvoir les principes du contrat d'engagement républicain. On en vient à se demander si les fédérations seront encore des outils au service d'une véritable politique sportive, ou si elles devront remplacer l'Observatoire de la laïcité, dont vous avez annoncé la suppression, peut-être parce que le travail remarquable qu'il accomplissait

même si la prise de conscience est assez tardive. Cet article définit les obligations qui pèsent sur les associations et les fédérations sportives au regard du contrat d'engagement républicain. Il précise les modalités d'octroi, de suspension et de retrait de l'agrément sportif et leurs implications juridiques.

Cet amendement a pour objet que les fédérations sportives veillent à ce que leurs adhérents ne manifestent pas leur appartenance religieuse de façon ostentatoire. Cette disposition n'est qu'un décalque de la loi de 2004 prohibant les signes d'appartenance religieuse ostentatoires dans les écoles, collèges et lycées publics. Les valeurs de la République se doivent aussi d'être respectées dans les lieux sportifs.

Mon amendement tend à préciser que le port de signes religieux ostensibles est interdit lorsqu'on participe à des événements sportifs et à des compétitions sportives organisées par les fédérations sportives et les associations affiliées. Il vise donc bien les compétitions nationales officielles organisées par les fédérations.

Dans son rapport, la commission d'enquête du Sénat sur les réponses apportées par les autorités publiques au développement de la radicalisation islamiste et les moyens de la combattre préconise d'introduire dans les statuts de chaque fédération sportive l'interdiction de toute propagande politique, religieuse ou raciale, telle qu'elle est prévue par la règle 50 de la Charte olympique. Notre pays accueillera les jeux Olympiques en 2024. Dans cette perspective, nous devons dès maintenant anticiper et préparer les fédérations sportives à respecter au plus vite les règles du Comité international olympique en matière de neutralité.

aucune sorte de démonstration ou de propagande politique, religieuse ou raciale n'est autorisée dans un lieu, site ou autre emplacement olympique Un terrain de football, un stade ou encore un gymnase sont des lieux qui doivent rester neutres, à l'abri de toute expression politique ou religieuse. Le sport véhicule des valeurs, en particulier celles d'égalité, de respect et de fraternité, qui ne peuvent être garanties que dans la sérénité et sans aucun sectarisme. En outre, les événements sportifs brassent beaucoup de monde, en particulier un public jeune qu'il faut préserver de toute influence. L'amendement n° 592

cela signifie, par exemple, que l'on condamne totalement le comportement de ces basketteurs américains qui ont posé un genou à terre, il y a quelques semaines, en réaction à un crime raciste.

L'article 25 prévoit, au travers d'une dizaine d'alinéas, de renforcer le contrôle de l'agrément des associations sportives, ce qui permettrait d'éviter certaines dérives dans le sport. Mais, en l'état, cet agrément ne sert presque à rien.

Au regard des enjeux inhérents au milieu sportif, il est important que toutes les associations organisant une pratique sportive soient soumises à l'agrément sport, notamment parce que cet agrément implique également le respect de l'intégrité physique des mineurs.

qui pourrait très certainement créer de fortes inégalités entre les associations sportives et les associations non sportives auxquelles aucun agrément n'est demandé pour solliciter et obtenir des subventions. L'agrément sportif n'est pas le seul en vigueur : on peut citer l'agrément jeunesse et éducation populaire, les associations agréées par le ministère de l'éducation nationale, ou les associations agréées pour la protection de l'environnement, par exemple.

pourrait-elle recevoir des subventions, alors qu'une association sportive non agréée ne le pourrait pas ? Il s'agit, à mon sens, d'une première source d'inégalités. En outre, rappelons que le texte issu des travaux de la commission prévoit déjà un accès aux équipements sportifs réservé uniquement aux associations agréées. Toutes les associations auront donc l'obligation de signer le contrat d'engagement républicain, en application de l'article 6 du présent projet de loi, pour pouvoir solliciter des subventions. Le texte prévoit donc déjà de limiter

C'est d'autant plus vrai quand on se rappelle la place particulière des associations sportives dans bon nombre de quartiers. Nous l'évoquions la semaine dernière lors du débat que nous avons dédié à la politique sportive : cette année de quasi-interruption du sport amateur a vu resurgir les effets néfastes l'on observait quand les associations sportives n'étaient plus sur le terrain- exclusion et déclassement social, mal-être, augmentation des risques psychologiques, occupation sauvage des lieux, etc. Bien entendu, il ne faut pas fermer les yeux sur certaines dérives qui peuvent apparaître, notamment dans certaines disciplines, comme le football et les arts martiaux. Le premier, sport qui regroupe le plus de licenciés dans le pays, constitue forcément une cible de choix. Les seconds ont été investis, comme les clubs de tir d'ailleurs, par des mouvements violents en quête d'entraînement. Toutefois, il faut faire

garanties doivent être réunies pour que la création du contrat d'engagement républicain ne conduise pas à la disparition d'associations tout à fait légitimes. Dès à présent, je note une différence avec l'article 6 : c'est un décret qui fixera les contours de ce contrat.

pour les fédérations agréées, d'organiser des actions de sensibilisation aux principes de la charte des engagements réciproques. Cette disposition nous interpelle à deux titres. Premièrement, le présent article prévoit déjà que le contrat d'engagement républicain comporte l'engagement, pour les fédérations agréées, de participer à la promotion et à la diffusion auprès des acteurs et publics de leur discipline des principes de la République détaillés dans ce contrat. Sur ce point, la précision apportée en commission paraît donc redondante. Deuxièmement et surtout, le renvoi à la charte des engagements réciproques était justifié par la volonté de conférer une base légale à ce texte, en lieu et place du contrat d'engagement républicain créé par ce projet de loi. Or le contrat d'engagement républicain a été pleinement approuvé et maintenu par les commissions des lois et de la culture, aussi bien à l'article 6 qu'à l'article 25. Ainsi, notre amendement vise à garantir la cohérence de cette disposition avec le projet de loi, tel qu'il résulte de son examen en commission. L'amendement

est favorable à l'amendement n° 593 rectifié : dans le cadre de la nouvelle répartition des rôles entre fédérations et État, les fédérations doivent prendre toute leur responsabilité afin de s'assurer, en leur sein, du respect du contrat d'engagement républicain et, plus généralement, de l'accomplissement des missions qui leur sont dévolues par l'État. Il s'agit également de mettre fin

Il tend à compléter l'amendement adopté lors de l'examen en commission, sur la proposition de M. le rapporteur pour avis, afin de prévoir un système d'agrément des associations sportives par les fédérations, seulement si l'association est affiliée à une fédération agréée.

Cet article impose une information régulière des élus concernés, par le préfet du département, quant à la situation des associations agréées dans leur territoire. Cette obligation nous semble très lourde

Il n'est pas opportun de prévoir, lors de la prise de licence, un contrôle, par les clubs [ ...]. » J'ai toujours compris que c'était aux fédérations

sur le contrôle d'honorabilité,

Il tend à mettre en cohérence la relation entre une fédération sportive délégataire et sa ligue professionnelle, afin de s'assurer du rôle de chacun des acteurs dans la mise en oeuvre de la stratégie nationale de la fédération concernée, visant à promouvoir les principes du contrat d'engagement républicain avec sa ligue. à garantir une implication plus large des ligues professionnelles dans la promotion des principes et des objectifs du contrat d'engagement républicain, conclu par les fédérations dans le cadre de leur agrément.

Le délai ainsi laissé paraît bien trop court, tant pour les fédérations que pour notre administration. Il existe aujourd'hui 115 fédérations sportives agréées par le ministère de la jeunesse

Cela est d'autant plus incohérent que les clubs sportifs verront leur agrément expirer dans un délai de trente-six mois après la promulgation de la présente loi, soit au mieux à la mi-2024. Il paraît étonnant que les agréments des fédérations sportives expirent avant

Comme je l'ai précisé dans mon propos introductif, le mouvement sportif a pleinement participé à l'élaboration du concept de contrats de délégation. C'est pourquoi il consent à ce

: cet amendement tend à étendre le contrôle d'honorabilité des encadrants des activités physiques.

aux établissements de premier et de second degrés. Je rappelle aussi que des obligations d'affichage existent déjà dans différents lieux, comme l'affichage des diplômes des intervenants, l'affichage de l'interdiction de fumer, l'affichage du 119,

qui ne se trouvent pas dans le cadre fédéral et échappent donc à tout contrôle. Ainsi, les établissements accueillant des activités physiques ou sportives devront assurer le respect des principes de la République, de la laïcité ainsi que l'interdiction de toute forme de prosélytisme religieux.

Dans de nombreuses communes, les équipements sportifs servent également de lieu d'accueil pour d'autres associations. Il convient donc de supprimer cet article, qui est un blanc-seing donné à ceux qui voudraient s'adonner à la partialité et régler leurs comptes avec une association qui leur serait opposée. Quel

présenter l'amendement n° 327. L'article 25 B, introduit en commission, réserve l'utilisation des équipements sportifs aux seules associations agréées. Il s'agit une nouvelle fois d'une mesure qui comporte plusieurs dangers et qui, surtout, ne répond à aucune demande des associations, ni même des collectivités. Ce dispositif exclurait de nombreuses associations non agréées qui, sans toucher de subventions de la part des collectivités, bénéficient de la mise à disposition d'un gymnase ou d'un stade. C'est notamment le cas de certains clubs sportifs loisirs. Le tissu associatif serait ainsi de nouveau fragilisé, alors qu'il n'est absolument pas démontré que le nouvel agrément soumis à la signature d'un contrat d'engagement républicain permettra de réduire les comportements communautaristes qui peuvent exister dans certains clubs.

Cessons d'alourdir les procédures pour les bénévoles associatifs. Nous vous proposons donc de supprimer cet article. La

Soyons honnêtes : la multiplication des associations sportives, accompagnée d'un manque d'équipement chronique, entraîne une réelle compétition pour les lieux. En pratique, les collectivités territoriales n'attribuent ces créneaux d'utilisation qu'à des associations agréées, sauf cas extrêmement rare. Le risque que des associations en bénéficient est donc particulièrement faible. En revanche, et c'est une réalité, il est fréquent que les collectivités, voire les clubs autorisent ou tolèrent la présence de pratiquants libres sur les équipements. Cela se fait soit en dehors des créneaux attribués, grâce à des créneaux libérés, soit dans une sorte de cohabitation. L'exemple le plus fréquent, c'est un centre d'entraînement composé de plusieurs terrains, dont un seul est occupé par un club, les deux ou trois autres étant libérés pour permettre à certains de jouer. Ce modèle d'occupation

de faire en sorte que le secteur sportif prenne toute sa place dans le renforcement du pacte républicain et la défense des principes de la République. la raison pour laquelle l'article 25 impose désormais aux fédérations sportives non seulement de signer le contrat d'engagement républicain, mais aussi, pour celles qui sollicitent une délégation de service public, de se doter d'une stratégie de promotion des principes de la République. Il a été introduit à l'Assemblée nationale que cette stratégie intègre des modules de formation obligatoires sur l'éducation aux valeurs et principes de la République. Nous défendons ces formations, mais l'alinéa dont nous proposons la suppression

: La parole est à M. Jean Bacci. Il s'agit d'un amendement de suite. Dans la mesure où il nous semble plus pertinent de faire reposer le contrôle des associations par l'État et les collectivités sur la charte des engagements réciproques, il est normal que nous amendions aussi cet article.

l'on nous propose d'inscrire dans le code de l'éducation. Je le cite : « L'organisation et l'enseignement de l'éducation physique et sportive participe à la promotion des valeurs de la République, notamment la liberté, l'égalité et la fraternité et se fait dans le strict respect de la laïcité. de la laïcité. » Mes chers collègues, c'est toute l'école de la République qui participe à la promotion des valeurs de la République, ce sont toutes les matières qui encouragent, en tout cas je l'espère, l'apprentissage des valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité, et ce sont tous les professeurs qui respectent le principe de laïcité

une. Mais laquelle ? Pour ce qui me concerne, la réponse est claire : il faut conserver la charte du Comité national olympique et sportif français et non celle de l'Agence nationale du sport. Pourquoi ? Ces deux structures sont de nature différente.

le même respect des principes de la République. Le CNOSF et le CPSF seront donc tout à fait dans leur rôle en indiquant la direction aux fédérations

reliée à l'État par une convention. Cette convention, que nous avons signée récemment, mentionne que toutes les subventions octroyées par l'ANS aux fédérations, aux associations sportives ou aux collectivités pour la construction d'équipements seront soumises

Lozach. Cet amendement tend à préciser que les concours de l'ANS aux différents projets et notamment à ceux des fédérations sportives se réaliseront dans le respect des principes du contrat d'engagements républicain. L'ANS pourrait ainsi soumettre le conventionnement des fédérations sportives au respect de ces principes.